tempérer le principe de liberté d'installation des médecins, notamment en passant par la négociation conventionnelle. Je vais m'efforcer, autant que faire se peut, de synthétiser et clarifier les termes du débat.

, 422 et 437 rectifié vise à préciser que le principe déontologique fondamental de la liberté d'installation des médecins, repris par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, doit être interprété au regard du principe d'égal accès aux soins. Je ne suis pas favorable à ce que cela figure dans la loi. L'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale fait référence à des principes déontologiques fondamentaux. Or le principe d'égal accès aux soins ne figure pas dans le code de déontologie médicale. Un second groupe d'amendements tend à encadrer l'installation des médecins par voie conventionnelle, selon des paramètres et des modalités distincts et, parfois, originaux. Une limitation de l'accès au conventionnement dans les zones surdenses est proposée par les amendements n 232 rectifié et 233 rectifié dans le second cas sous la forme d'une expérimentation.

à la négociation conventionnelle pour la mise en place de mesures restrictives au conventionnement en zones surdenses, et, dans un second temps, en cas d'absence de négociation sur ce thème dans les douze mois, l'application d'un dispositif restrictif à l'accès au conventionnement dans ces zones. Selon les amendements, l'application de ce dispositif supplétif se fait, ou non, de manière expérimentale. Deux autres amendements identiques- les

des conditions limitatives d'accès au conventionnement en d'autres points du territoire. La commission n'est pas favorable à la définition de mesures restrictives au conventionnement, ne serait-ce qu'en raison de leur faible efficacité en pratique, voire de leur caractère contre-productif. Plusieurs professions de santé ont mis en place un conventionnement collectif. Dans certains territoires, il en a résulté d'importants effets de seuil les professionnels s'installent à la marge des zones sous-denses, tout en exerçant dans d'autres zones. Certains pays comme l'Allemagne et le Canada ont également développé des mesures de conventionnement sélectif. Cela a favorisé l'éclosion d'une médecine à deux vitesses à grande échelle, de nombreux praticiens ayant décidé de se conventionner auprès d'assurances privées.

elle fait un pas symbolique, tout en laissant une large marge de manoeuvre aux partenaires conventionnels. Cette rédaction est, par ailleurs, proche de celle que le Sénat avait adoptée à l'article 12 A du dernier projet de loi

visent à restreindre la liberté d'installation. Je le répète, seulement 5 % des jeunes médecins veulent s'installer. Nous pouvons en être certains, si l'on restreint encore plus la liberté d'installation,

les médecins généralistes doivent être formés à la gynécologie médicale, et les sages-femmes ont le droit de faire des frottis et de suivre les grossesses non pathologiques des femmes. Ainsi convient-il de mieux répartir la tâche entre d'autres professionnels, en attendant que des gynécologues médicaux sortent des facultés.

À l'inverse, dans les CPTS, le collectif de professionnels de santé s'engagera sur une responsabilité de type. Le cahier des charges a été négocié dans la convention médicale ; il vise à garantir

pour réguler l'installation des médecins sur notre territoire et lutter contre les déserts médicaux. Il faut par exemple lutter contre le recul des services publics. En effet, aucun médecin n'acceptera volontiers de s'installer dans une zone rurale qui a vu

les enseignants nommés dans un endroit qui ne leur plaît pas feraient de l'enseignement de mauvaise qualité. Et les gendarmes et les policiers nommés là où ils ne veulent pas aller feraient de la police de mauvaise qualité. Un tel raisonnement

L'Allemagne a inscrit dans sa loi fondamentale le principe de la liberté d'exercice et d'établissement. Pourtant, cela n'a pas empêché le législateur allemand de restreindre fortement la liberté d'installation, au nom de l'égal accès aux soins,

où la désertification n'est pas une idée en l'air, mais une réalité. Dans un département rural comme le mien, la Dordogne, nous avons des cantons qui n'ont plus de médecins. Vous nous dites, madame la ministre, qu'avant vous d'autres ministres de sensibilités différentes ont eu la même réaction devant de telles propositions, qui émanaient notamment

a déroulé le tapis rouge, ou presque. Résultat : la réalité, sur le terrain, continue de nous interpeller. Il est plus que temps de réagir et de remédier à ce problème que sont les déserts médicaux. C'est un fait : la répartition des médecins n'est pas équitable sur le territoire. Cela ne pose-t-il pas un grave problème de santé publique ? Dans mon

rien à redire. Madame la ministre, nous avons été plusieurs à déposer des amendements que vous avez refusés d'un revers de main ; il s'agissait d'imaginer de quelle manière on pouvait encourager les médecins à s'installer sur des territoires en déprise. Aujourd'hui, vous refusez des amendements

cette insuffisante professionnalisation de la formation est à l'origine du délai très important entre la fin des études et l'installation. Vous présentez un projet de loi qui contient un chapitre dédié à la formation,

! Comment peut-on travailler dans ces conditions ? Vous nous mettez dans une situation impossible. Madame la ministre, je vous le dis très tranquillement : je serais ravi si l'adoption du projet de loi que vous nous présentez fait que, dans quatre ou cinq ans, le problème est à peu près réglé. Mais il ne le sera pas ! Il le sera à l'échéance de l'évolution de la démographie médicale ; mais l'impulsion que vous donnez est tout à fait insuffisante. Je voterai- nous voterons -l'amendement de la commission du développement durable, mais ce débat ne sera évidemment pas clos. Et s'il ne l'est pas, c'est à cause de votre incapacité à écouter et à nous proposer des mesures plus volontaristes.

Vous confirmez que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a donné aucun résultat ; et évidemment, cela a été dit, votre plaidoirie se retourne contre vous, parce que vous ne proposez rien. Vous

le Royaume-Uni également ; l'Allemagne se lance aussi dans ce conventionnement sélectif, comme les Pays-Bas. Les pays d'Europe ont les mêmes problèmes que nous.

C'est donc bien l'absence de contrainte à l'installation, et elle seule, qui explique le problème des déserts médicaux. Si ce problème est plus important en France, c'est justement parce que nous n'avons aucune contrainte.

Mais, madame la ministre, si vous voulez, je vous trouve un rendez-vous chez un spécialiste, dans le quartier, dans moins d'une semaine ! Hier, j'ai rencontré un maire qui, dans mon département, avait obtenu un rendez-vous chez un ophtalmologue ... en février prochain.

que l'Allemagne a dû constater que la régulation était un échec, c'est totalement faux, ... Totalement ! ... et vous le savez très bien, puisque, très récemment, très récemment, le 6 mai 2019- ce n'est pas ancien ! -, les Allemands ont voté une loi qui confirme la régulation et qui donne simplement un peu plus de pouvoir aux régions.

Il y a là un enjeu d'égal accès à la santé ; c'est particulièrement sensible dans des départements où l'état sanitaire de la population est médiocre, voire mauvais. aggrave l'enjeu de l'accès de ces populations à des médecins qui doivent être en nombre suffisant, et légitime encore un peu plus cette régulation attendue par tous. Il y va de la responsabilité des autorités politiques en charge de la santé- les Français sauront apprécier. Il y va éventuellement de leur responsabilité judiciaire, qui, un jour ou l'autre, ne manquera pas d'être engagée.

oeuvre de contrats locaux de santé. Je puis vous citer des territoires qui en sont déjà à leur troisième contrat local de santé ; ils ont pu ainsi créer une véritable dynamique et intéresser de nouveaux professionnels de santé.

explication de vote. Notre collègue Élisabeth Doineau a eu raison de rappeler qu'il n'y avait pas de solution miracle à la situation que connaissent les territoires. Il n'empêche que nous avons une obligation

Madame la ministre, je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par vos arguments. Vous avez cité un certain nombre de professions de santé : les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les sages-femmes, en précisant que ces professions étaient surdotées. Il y en a une que vous n'avez pas citée

serait rude. Je le vois depuis le premier jour dans tous mes déplacements : elle est terriblement rude. La douleur dans les territoires, vous n'êtes pas les seuls à la sentir ; vous n'êtes pas les seuls témoins des territoires. Chacun d'entre nous a des liens ou de la famille dans tous les territoires de France. Très bien ! Je pense depuis le premier jour qu'il y a urgence à agir. Depuis le mois de juin 2017, je travaille sur un plan d'urgence d'accès aux soins. Celui-ci a été annoncé. Il contient des mesures facilitatrices pour l'installation des médecins, pour le cumul emploi-retraite, pour créer des postes d'assistants salariés, des postes d'assistants spécialisés dans les outre-mer. Il a été présenté par le Premier ministre au mois d'octobre 2017. J'ai souhaité ensuite aller vers une transformation beaucoup plus globale, utilisant tous les leviers possibles : la formation, le financement de la médecine, le numérique, l'organisation. J'ai fait travailler des gens pendant un an. Le résultat, c'est ce texte.

Beaucoup d'entre vous me disent que cela ne suffit pas et n'a pas marché. Mais si cela n'a pas marché, c'est parce que, jusqu'à présent, on a pensé le modèle

et M. Amiel l'ont souligné. Il n'est pas bien de dire que les médecins n'ont pas de prise de conscience ! Tous les professionnels de santé ont pris conscience de la nécessité de transformer le système. Ils sont engagés

Par ailleurs, les jeunes sont engagés. Ils sont remarquablement raisonnables. Ils ont un sens du service public. Ils ont un sens de la santé publique et de la prévention. Mais ils nous disent qu'ils veulent exercer

un peu plus loin ! Ne dites pas que je ne prends pas mes responsabilités. Je les prends complètement. Je me sens responsable de la santé des Français. Sinon, je ne serais pas là. Je veux terminer par une très belle citation de Nelson Mandela,

Le scrutin est ouvert.

le dîner -tendent à insérer dans le code de la sécurité publique, après les mots « liberté d'installation du médecin », les mots « sans préjudice du respect du principe d'égal accès aux soins ». Il ne s'agit pas d'une mesure de coercition.

Le scrutin est ouvert.

commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

et les médecins libéraux. Ces rapports seraient définis par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le Conseil national de l'ordre des médecins, et non les syndicats.

Le scrutin est ouvert.

... Il s'agit ici de conditionner le conventionnement des médecins avec l'assurance maladie à leur installation dans un délai raisonnable après la soutenance de leur thèse.

Ces médecins bénéficieraient d'un statut propre qui ne se confondrait ni avec celui des médecins remplaçants, puisque les médecins qu'ils viendraient épauler ne cesseraient pas leur activité, ni avec celui des médecins adjoints, puisque les médecins venant en renfort exerceraient pour leur propre compte. Ce statut permettrait notamment de limiter le poids des charges sociales et de soumettre ces médecins à un régime d'assurance maladie aligné sur celui des salariés.

Plusieurs outils existent déjà pour permettre l'exercice ponctuel de la médecine dans certains territoires et dans certaines situations qui le nécessitent ; je pense aux statuts de médecin remplaçant, de médecin adjoint, pour les médecins non thésés, et de médecin assistant, pour les praticiens diplômés. Il n'a pas paru opportun à la commission de complexifier encore ces outils, leur paysage étant déjà peu lisible, si j'en crois les discussions que nous avons eues à ce sujet.

Actuellement, les médecins peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales au titre de l'embauche d'un salarié, mais également de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, au titre d'une installation dans une zone de revitalisation

collègues, ce n'est vraiment pas d'une grande efficacité ... Si l'on veut faire évoluer notre système de protection sociale, cette ambition doit s'appuyer sur un financement à la hauteur des besoins en santé de notre siècle

Estrosi Sassone. Cet amendement a pour objet de rendre encore plus attractive l'installation de médecins dans les territoires sous-dotés, en ajoutant à l'exonération des cotisations sociales celle de l'impôt sur les bénéfices pendant les cinq ans suivant leur installation.

n'avaient jamais fait l'objet d'évaluation, malgré la multiplication, au cours des dernières années, des aides de l'État et des collectivités s'ajoutant à des dispositifs conventionnels. Elle avait aussi constaté que ces aides n'avaient pas enrayé l'accroissement des inégalités territoriales dans l'accès aux soins, comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises et comme la commission l'a rappelé dans ses travaux. Il est donc permis d'avoir des doutes quant à l'efficacité de ces dispositifs, de surcroît coûteux pour les finances publiques. La Cour des comptes a ainsi estimé que, pour le seul périmètre de l'État et de l'assurance maladie, ces dispositifs représentaient, en 2015, près de 90 millions d'euros. Dans une démarche de compromis, notre commission propose donc un meilleur ciblage du dispositif, afin de rendre celui-ci plus efficace en le concentrant sur les territoires qui en ont le plus besoin. Pour limiter son impact sur les finances publiques, cette mesure doit être comprise en miroir et en cohérence avec les autres mesures que nous avons proposées pour améliorer l'accès aux soins. La parole

semble que l'ensemble du dispositif va dans le sens de M. Longeot. Ce sous-amendement vise à cibler davantage le mécanisme d'exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins, proposé à l'article 4 , sur les zones sous-médicalisées. Il s'agit ainsi d'encourager plus efficacement l'installation des jeunes médecins dans les déserts médicaux, en concentrant les incitations sur les territoires carencés en médecins tout en limitant l'incidence

proposé octroie une exonération fiscale aux médecins retraités. Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, afin d'encourager les médecins à prolonger leur exercice.

Il s'agit d'une mesure de bon sens qui permet d'apporter une première réponse d'urgence aux problèmes de démographie médicale. Ce dispositif instaure une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin installé ou à la recherche d'une installation en exercice libéral.

de l'amendement, il leur reviendrait en effet de proposer la création de zones franches médicales -et sur les conditions dans lesquelles des médecins retraités s'installeraient, sachant qu'une réinstallation d'un praticien préalablement installé n'est pas considérée comme une nouvelle installation.

Cette proportion paraît d'autant moins déraisonnable que le remplacement répond à un besoin véritable des acteurs du système de santé. Le recours à des remplaçants est en effet essentiel pour assurer la continuité des soins, notamment lorsqu'un médecin prend ses congés. Une diminution du vivier de remplaçants risquerait, dans ce contexte, de laisser des territoires sans médecins pendant plusieurs semaines, chaque année, durant des périodes critiques comme l'été. Cette diminution pourrait également dégrader le confort d'exercice des médecins, particulièrement dans les territoires les plus fragiles, en limitant leurs possibilités de s'absenter pour motifs personnels ou pour suivre des formations. Les territoires fragiles, qui peinent à attirer des médecins remplaçants, seraient les premiers à subir les effets de cette dégradation. Par ailleurs, un médecin qui changerait de situation- en cas de déménagement, par exemple -pourrait se voir interdire de remplacer durant l'intervalle entre deux installations, ce qui limiterait d'autant le temps médical disponible pour la population. L'exercice, en tant que remplaçant, permet aussi aux jeunes médecins de réfléchir à leur projet professionnel et de préparer leur installation : 81 % des installés ont d'abord été remplaçants exclusifs, selon une récente étude du Conseil de l'ordre. Restreindre cette possibilité risquerait de dégrader encore l'attractivité l'attractivité de l'exercice libéral et, à l'inverse, de renforcer l'attrait du salariat. Enfin, il me semble que cet article pose un problème au regard du principe d'égalité, notamment entre les médecins de plein exercice, pour lesquels on érigerait une limite dans le temps à leur capacité de remplacer, et les futurs médecins ayant une autorisation de remplacement qui resterait sans limite. La question de la constitutionnalité d'une telle différence de traitement peut donc se poser. Le Gouvernement entend privilégier une politique d'accompagnement des débuts d'exercice en libéral. dans sa rédaction actuelle, cet article va à l'encontre de cette dynamique d'installation. Une telle disposition devrait être travaillée de concert avec les représentants des professionnels concernés

Si l'article 4 était maintenu, on risquerait de voir des jeunes mal préparés à l'installation ou n'ayant pas envie de s'installer tout de suite se réfugier vers la pratique hospitalière et salariée, ce qui irait à l'inverse de ce que nous voulons tous, à savoir davantage d'installations en ambulatoire.

Je comprends parfaitement la démarche du rapporteur, dans ces temps d'urgence, tendant à accélérer l'installation d'un millier de jeunes médecins supplémentaires. Aujourd'hui, notre système de santé est en grande difficulté et a grand besoin d'être réformé. nous accordons tous sur ce point. Mais céder aux sirènes trompeuses de la coercition ne fera qu'achever la médecine libérale. Les jeunes médecins ne doivent pas être une variable d'ajustement des erreurs du passé. Beaucoup d'entre eux, c'est vrai, font des remplacements durant leurs premières années d'exercice, mais on ne peut pas penser sincèrement et sérieusement, mes chers collègues, que c'est au détriment des patients et du maillage territorial que nous appelons tous de tous de nos voeux. Les médecins remplaçants répondent à un véritable besoin de santé ; ils assurent la continuité de l'accès aux soins dans nos territoires, parce que les médecins qu'ils remplacent prennent quelques congés ou consacrent du temps à leur formation continue. Il est indispensable d'inciter les jeunes professionnels à l'installation, mais nous ne pouvons pas le faire en les emprisonnant dans de fausses alternatives : ce ne sont pas des pions sur l'échiquier des territoires. Je vous le dis, mes chers collègues : notre responsabilité de législateur ne peut pas être de céder aux pressions des fossoyeurs de l'exercice libéral, dont l'idéal de fonctionnarisation de la médecine pour enrayer la désertification médicale n'est qu'une chimère. La redynamisation sanitaire de nos territoires ne pourra se faire contre les médecins. Faisons-leur confiance et laissons-les libres sur le terrain de leur installation et de leur mode d'exercice. La parole est à Mme Laurence Cohen,

J'avoue que je suis un peu surprise de la tournure que prend cette discussion : certains collègues n'ont jamais de mots assez forts pour défendre la liberté d'installation ; et là, tout d'un coup, de liberté, il ne pourrait plus être question ! Nous avons et nous aurons toujours besoin de médecins remplaçants, jeunes ou moins jeunes. J'ai J'ai la chance de vivre dans un département côtier qui compte des stations touristiques ayant besoin de médecins à certaines périodes de l'année plus qu'à d'autres- c'est le cas aussi dans les zones montagneuses.

deux médecins d'une même maison de santé pluriprofessionnelle : quand l'un part en vacances, l'autre récupère la patientèle et perçoit une rétrocession sur l'activité. En réalité, le remplacement est un mode d'exercice sur le terrain. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est médecin remplaçant, on n'est pas en activité.

merci.